de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le problème, c'est la chute des effectifs de la DGCCRF, avec la fermeture des directions départementales où le nombre d'agents s'était réduit, et l'insuffisance notable de moyens humains sur certains dossiers

Le déclin du service public de l'État pose évidemment de grandes questions pour ce qui relève de la sécurité alimentaire, des capacités d'investigation de l'Autorité de la concurrence et du caractère uniquement facultatif d'un certain nombre de ses décisions.

et le taux de concentration atteignait 80 %. Aujourd'hui, celui-ci est égal à 90 %, et on nous annonce la fusion des centrales d'achat de Casino, Auchan et Système U. Nous sommes face à un système d'oligopole qui tue notre économie agricole en confisquant la valeur ajoutée. Malgré les textes législatifs successifs, rien n'est fait contre ce système de concentration toujours plus poussée de la grande distribution. de la concurrence a estimé que les accords de coopération permettant cette concentration n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle préalable au titre des concentrations et ne pouvaient être examinés qu'au regard du droit des ententes anti-concurrentielles. Certes, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a institué une obligation de communication préalable à l'Autorité de la concurrence des accords de rapprochement à l'achat, mais cela n'est manifestement pas suffisant. Pourtant, c'est bien à cause de ce système que 30 % de nos agriculteurs gagnent aujourd'hui moins de 350 euros par mois Aussi, nous vous proposons de compléter la procédure permettant à l'Autorité de la concurrence d'évaluer l'effet anti-concurrentiel de la mise en oeuvre des accords de coopération à l'achat entre enseignes de la grande distribution de produits alimentaires. Il est ainsi proposé

En effet, la loi ne doit pas laisser envisager que des atteintes à la concurrence soient admises. L'important réside dans la caractérisation des impacts économiques sur les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. rendre systématique l'intervention de l'Autorité de la concurrence pour la mise en oeuvre de mesures conservatoires, si elle a constaté des atteintes à la concurrence ou sur les différents maillons de la chaîne. rendre publics le bilan concurrentiel ainsi que les engagements pris par les parties et d'expliciter dans quel cas l'Autorité de la concurrence prend des mesures conservatoires. C'est tout le sens de cet amendement auquel, j'en suis sûr, M. le ministre sera favorable. L'amendement

au même titre que le ministre de l'économie, à demander à l'Autorité de la concurrence de réaliser le bilan concurrentiel de mise en oeuvre des accords de regroupement prévu à cet article. Nous estimons que les parlementaires ont un rôle de lanceur d'alerte à jouer et doivent être en mesure, lorsque des informations concordantes semblent indiquer la constitution d'un oligopole, de consulter l'Autorité de la concurrence. À l'Assemblée nationale, vous avez indiqué, monsieur le ministre, que le Parlement ne pouvait pas saisir l'Autorité de la concurrence. Nous estimons nécessaire, dans ce cas,

Henri Cabanel. L'alinéa 9 de l'article 10 A dispose que l'Autorité de la concurrence apprécie si l'accord de rapprochement apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence. nous estimons que l'Autorité de la concurrence doit intégrer dans sa réflexion une dimension sociale et qualitative. Le seul élément économique n'est pas suffisant, et les dérives que nous connaissons actuellement en France avec la concentration des centrales d'achat en sont une illustration.

publics. Si nous pouvons considérer que cet article constitue une petite avancée en matière de lutte contre certains accords de coopération dommageables, nous regrettons que l'action de l'Autorité de la concurrence survienne après les rapprochements. Dans ce cadre, même si l'Autorité de la concurrence pourra demander la prise de certaines mesures en cas d'atteinte à la concurrence, nous nous interrogeons sur la réelle effectivité de son action. Pour autant- ce fut rappelé à maintes reprises lors des débats à l'Assemblée nationale comme en commission au Sénat -, nous serions allés ici au maximum de ce qu'autorise la réglementation européenne. C'est pourquoi nous proposons que les bilans concurrentiels de l'Autorité de la concurrence ainsi que ses recommandations soient rendus publics. En effet, le texte actuel prévoit que l'engagement de la procédure est rendu public, mais rien n'est indiqué quant aux conclusions.

Il n'est pas sûr que ce soit le rôle du Parlement de solliciter une saisine dans un dossier individuel. Cet amendement tend également à préciser que le bilan se fait au regard de la création ou du renforcement d'une position dominante.

aussi à rendre publics le bilan concurrentiel et les engagements. Afin de respecter le secret des affaires, il ne paraît pas souhaitable de publier le bilan concurrentiel et les engagements des parties dans leur totalité. Bien évidemment, cela n'empêchera pas l'Autorité par voie de communiqué de presse, comme elle le fait couramment, de faire état de ses constatations et des engagements pris par les intervenants. est inutile de rendre systématique la prise de mesures conservatoires. Le dispositif proposé par l'article 10 A semble suffisant pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'intervenir, selon un principe de proportionnalité qui s'applique à ses décisions.

déjà saisir l'Autorité de la concurrence pour avis pour toute question relative à la concurrence, indépendamment d'une procédure d'examen en cours. Il est par ailleurs informé des activités de l'Autorité de la concurrence chaque année. Il n'est sans doute pas souhaitable d'aller au-delà. La commission a émis un avis défavorable sur

Ainsi, l'article L. 420-4 du code de commerce exclut l'interdiction des ententes ou des abus de position dominante lorsqu'ils se traduisent par un progrès pour l'emploi.

est vrai que l'Autorité de la concurrence peut avoir recours aux effectifs de la DGCCRF, de même que la DGCCRF peut transmettre à l'Autorité de la concurrence des indices de pratiques anti-concurrentielles. Ce faisant, il s'agit d'accroître l'efficacité de leurs actions respectives. Aujourd'hui, la DGCCRF compte à peu près 3 000 agents

car elle permet de contrôler l'ensemble des accords en cours. Le contrôle, qui est mis en place, nous permettra d'aller, si nécessaire, jusqu'à l'interdiction des accords, si le bilan concurrentiel révèle des pratiques illicites.

Monsieur Bérit-Débat,

qui soulève la question de la dépendance économique des producteurs vis-à-vis des acheteurs. Nous ne pouvons le nier : de nombreux producteurs sont aujourd'hui pieds et poings liés face à leur distributeur. Il convient une nouvelle fois de mieux protéger les plus faibles parties du contrat, à savoir les exploitants, dans la relation commerciale. Caractériser de façon améliorative la dépendance économique, c'est faciliter les poursuites dans le contexte le contexte de création d'un groupement de grandes enseignes de la distribution, capables de faire pression sur l'ensemble des acteurs se situant en amont de la chaîne de vente et d'imposer des conditions défavorables aux agriculteurs. Il paraît inacceptable qu'agriculteurs ou fournisseurs de la grande distribution puissent être soumis à un tel déséquilibre, qui les laisse parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables. Quel

cet amendement est bien nécessaire, compte tenu de l'amélioration des dispositifs de répression des comportements abusifs et restrictifs de concurrence qui devraient résulter de l'ordonnance qui sera prise sur la base de l'article 10 de ce projet de loi. En outre, sur le fond-

un impact plus défavorable qu'aujourd'hui pour les petites et moyennes entreprises, en poussant les distributeurs à des comportements « malthusiens » qui auraient pour seul but de les protéger juridiquement contre la mise en jeu de leur responsabilité dans le cadre de relations commerciales qu'ils auraient nouées qu'ils auraient nouées avec des fournisseurs qui sont des PME. Potentiellement, le risque est que les distributeurs privilégient des grands groupes qui n'auront pas un lien de dépendance « structurelle » avec eux, contrairement à certaines PME. Par conséquent, l'avis est défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

proportionné aux avantages qui sont tirés du manquement à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques. Dans ces conditions, puisqu'un dispositif

Cet amendement, qui nous a notamment été proposé par le syndicat majoritaire, vise à répondre à la problématique de la concentration toujours plus importante des centrales d'achat, que nous avons déjà évoquée. Ces rapprochements ont été permis par l'Autorité de la concurrence française, qui les considère comme des « accords de coopération comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Or la concentration excessive des centrales d'achat de la grande distribution met en péril l'équilibre même des négociations commerciales, créant de nombreuses situations de dépendance économique. Il est impératif de mettre un terme à ce système qui est à bout de souffle, voire qui n'a jamais fonctionné et qui ne sert personne. Agriculteurs, PME, entreprises de taille intermédiaire, consommateurs, salariés : personne n'est épargné. n'est épargné. Afin d'éviter que ce type de rapprochement n'ait à nouveau lieu, il est nécessaire de prévoir que ce type d'accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l'Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l'accord : l'analyse de l'impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l'analyse de l'impact sur le consommateur.

C'est précisément compte tenu de cette situation qu'a été créé l'article L. 462-10 du code de commerce, qui prévoit depuis 2015 la transmission préalable de tels accords à l'Autorité de la concurrence et qui, en vertu de l'article 10 10 A, permettra d'assurer un bilan concurrentiel permettant de sanctionner les pratiques abusives dans ce domaine. L'extension du dispositif de contrôle des concentrations serait donc aujourd'hui inutile. Du reste,

d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence ». Ces pratiques peuvent consister aujourd'hui à organiser, pour les produits agricoles

Il tend à reconnaître les groupements d'agriculteurs, comme les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, les centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, les CIVAM, et les groupes d'étude et de développement agricole, notamment. Ces collectifs d'agriculteurs sont essentiels au lien social dans le monde rural. À l'heure où l'isolement et le repli sur soi gagnent de plus en plus d'agriculteurs en difficulté, où la concentration des fermes conduit à vider les campagnes, rappeler leur rôle. Ces collectifs permettent également une intégration dans le milieu agricole des nouveaux agriculteurs. Cette intégration est essentielle à l'heure où de plus en plus d'installations se font hors cadre familial.

nous devons leur donner toutes les chances de réussir à s'approprier ce beau métier d'agriculteur, souvent passionnant, mais aussi éminemment complexe. L'agriculture de groupe

notamment la transition écologique. En favorisant l'échange de pratiques, la réflexion collective, parfois en lien avec des chercheurs, ils permettent de trouver des solutions réellement efficaces, utiles aux paysans et à leur autonomie,

a une véritable portée juridique, essentielle pour favoriser la transition agricole. La parole

les GIEE, ou les CIVAM permettent aujourd'hui à des agriculteurs de se réunir pour être plus forts et plus efficaces. Ces collectifs sont des lieux d'innovation, d'entraide, de solidarité et, par là même, de lutte contre l'exclusion sociale et économique. Cela fait

« collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances, ainsi que de ressources humaines et matérielles

mais ce ne serait pas la première fois, mes chers collègues, que nous adopterions un amendement dont la dimension symbolique fait sens politique, dans l'intérêt de notre société.

en leur ouvrant la possibilité d'acquérir du foncier. C'est à ce moment que les agriculteurs, pour pouvoir s'organiser, ont commencé

territoire, une agriculture de résilience, dans laquelle le collectif retrouve toute sa force, en réponse à un individualisme exacerbé qui mène une partie de nos agriculteurs dans l'impasse.

ces amendements, il s'agit de réaffirmer l'importance de l'agriculture de groupe sous toutes ses formes, en lui donnant la reconnaissance législative dont elle a besoin.

En effet, le collectif, véritable levier de triple performance pour l'agriculture, doit être identifiable au travers d'une personne morale qui, de ce fait, peut incarner l'intérêt collectif de ses membres, permettre de renforcer la pérennité et la structuration du projet porté par les adhérents du collectif, réguler le fonctionnement entre agriculteurs parties prenantes par des règles juridiquement établies.

en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière, notamment en matière de contractualisation et de niveau de partage de la valeur. L'accord interprofessionnel en vigueur expirera le 30 septembre 2020. Les négociations relatives à l'accord interprofessionnel pour les récoltes de 2020 et au-delà commenceront donc au début de 2019 et devront se conclure avant la fin de la même année, soit avant la définition des assolements pour la campagne 2020-2021. Le rapport que nous demandons est d'une importance majeure pour conclure l'accord interprofessionnel le plus équilibré et le plus équitable possible.

l'avis du Gouvernement ? Cette demande de rapport a été adoptée à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement- ce sont des choses qui arrivent ! Depuis lors, je n'ai pas changé d'avis

la taxation à taux réduit avait été accordée pour les aliments de consommation courante, du fait de l'importance du budget alimentaire pour les ménages. À l'inverse, quelques aliments considérés comme des produits de luxe étaient taxés à taux plein. taux plein. Cette distinction est devenue obsolète du fait à la fois de l'amélioration du niveau de vie et de la banalisation de certains produits précédemment considérés comme luxueux. En revanche, une autre problématique est apparue : la surconsommation d'aliments transformés très gras ou très sucrés, qui se sont progressivement substitués à une alimentation plus saine.

quant aux adultes français, ils sont 49 % à être obèses ou en surpoids. Dans ce contexte d'une progression des habitudes alimentaires néfastes pour la santé et, de manière plus générale,

une reclassification des taux de TVA en fonction non seulement de l'intérêt nutritionnel des produits alimentaires, mais aussi de l'intérêt sanitaire et environnemental des produits de consommation courante.

Les auteurs de cet amendement proposent la remise au Gouvernement d'un rapport de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la reclassification des taux de TVA en fonction de l'intérêt nutritionnel, sanitaire et environnemental Une classification différenciée existe déjà dans le système français de TVA. Ainsi, les aliments de consommation courante sont soumis à un taux réduit, tandis que les aliments de luxe sont taxés à taux plein. Dans un contexte de progression de l'obésité, il pourrait être intéressant de réfléchir à une reclassification des taux de TVA en fonction de la qualité nutritionnelle, sanitaire et environnementale des aliments.

collègues sont au travail dans leur département

M. Franck Montaugé, sur l'article. Le rapport que prévoit cet article permettrait d'améliorer le dialogue et les échanges entre le Gouvernement et le Parlement, à un moment particulier où la Commission européenne annonce de profondes mutations des mécanismes de la politique agricole commune. mécanismes se traduiront par davantage de subsidiarité en matière d'atteinte des objectifs contractuels définis entre les États membres et la Commission européenne. Le rapport demandé permettrait aux commissions des affaires économiques et des affaires européennes des deux chambres d'exercer de manière plus efficiente leurs missions de contrôle et d'évaluation des politiques publiques- agricole en l'occurrence. Dans une première étape, en 2019, ce rapport permettrait au Gouvernement d'exposer et de soumettre à la réflexion du Parlement les orientations stratégiques qu'il entend faire prévaloir

PAC annoncée par les commissaires Oettinger et Hogan doit être anticipée du point de vue de ses conséquences directes et immédiates sur le revenu des agriculteurs : le risque d'une perte instantanée de la valeur hypothétiquement regagnée en améliorant les relations commerciales

et le plan d'action du Gouvernement pour préserver le potentiel d'innovation et de développement de nos agricultures, tout en répondant aux attentes de nos concitoyens en matière de qualité alimentaire.

tels que le CETA aura, nous le savons, des effets particulièrement désastreux sur notre agriculture. Il est essentiel que le Gouvernement rende des comptes au Parlement sur les engagements pris par la France dans ce contexte. De plus, la réforme de la PAC aura une influence cruciale sur notre agriculture. Le Sénat a souligné à de nombreuses reprises le risque de baisse du budget de la PAC et d'une renationalisation qui serait source de distorsions

La rémunération des services environnementaux était l'un des axes du discours de Rungis du Président de la République. Vous avez également annoncé qu'elle serait l'un des axes de la position que défendra la France dans le cadre des négociations sur la PAC. Or nous ne savons toujours pas quelles réalités vous mettez dernière ces termes, ni quelle vision vous défendez auprès de l'Union européenne. En parallèle, vous avez supprimé le financement national de l'aide au maintien en agriculture biologique, ... C'est faux ! ... que l'on pouvait considérer comme une rémunération des externalités positives liées à ce mode de production, en expliquant que le marché pouvait rémunérer l'agriculture biologique.

S'il doit y avoir mobilisation des parlementaires nationaux dans le cadre de la renégociation en cours de la PAC, cela doit être selon un mandat clair, avec des objectifs précis.

Au moment où s'ouvre le débat sur la réforme institutionnelle, la question de l'échange d'une information fiable et de qualité entre Gouvernement et Parlement n'est pas anodine. n'est pas anodine. Ces demandes fréquentes de rapports, trop souvent rejetées, devraient être reconsidérées à l'aune de l'efficacité de nos institutions, dans l'intérêt de la démocratie et de la République. C'est en tout cas ce que je pense.

européenne. Si je puis me permettre de donner un conseil à un ministre, appuyez-vous sur l'opinion publique nationale et européenne. On est en train de travailler à la création d'une opinion publique européenne

En effet, la surtransposition est l'une des maladies du droit français, ... Tout à fait ! ... tout spécialement en matière agricole et alimentaire. Cette pratique met en cause la compétitivité de nos filières agricoles et alimentaires. Transposer strictement les dispositifs communautaires n'implique aucunement une baisse de la qualité de nos productions. L'objet de cet amendement est donc de faire de la non-surtransposition et de la stricte proportionnalité dans la mise en oeuvre en droit français des règles européennes et internationales l'un des principes de notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation.

Dans une lettre en date du 11 juin dernier adressée au député européen Éric Andrieu, le commissaire européen à l'agriculture, M. Hogan, indique que « ses services ont expliqué aux autorités françaises les possibilités d'indexer le versement des aides aux contraintes et aux conditions d'exploitation agricole Dans mon département du Gers- mais je pourrais tout autant citer celui de l'Aude, cher à Gisèle Jourda -, il reste 109 exploitations dans des zones de coteaux où il n'est possible de faire que de l'élevage.

En conséquence, pour préserver cette aide essentielle au maintien de ces élevages et à la vie dans les territoires concernés, nous vous demandons de faire réaliser par vos services, dans le cadre des possibilités laissées par les règlements européens, en vue du classement des communes de ces territoires en zone intermédiaire de type piémont, par exemple, et de rendre publics les calculs détaillés justifiant la carte que vous soumettez à l'Union européenne, et ce pour chaque département de France.

placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Il a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution, ainsi que la répartition de la valeur ajoutée dans l'ensemble de la chaîne

SNBC, qui traduit concrètement les engagements pris par la France lors de la COP21. En effet, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation est à l'origine d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France. Ainsi, la transformation de notre production agricole et de notre alimentation est nécessaire, en particulier, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.

La SNBC indique également que le programme national relatif à la nutrition et à la santé devra intégrer les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dès sa révision, qui est en cours.

Il s'agit non pas de supprimer la viande, mais de privilégier la qualité, dans l'intérêt des éleveurs. Cet amendement vise à inscrire cette orientation dans le code de la santé publique. De plus, il tend à faire de l'éducation à l'alimentation et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques qui sous-tendent l'alimentation un levier de cette nécessaire transition.

contre les changements climatiques dans nos modes de production et de transformation. Améliorer la qualité de l'offre, c'est l'améliorer sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan environnemental. L'inscription de ces nouveaux objectifs dans le texte serait un signal très fort. L'amendement

Cet amendement vise à mettre le programme national pour l'alimentation en cohérence avec les objectifs de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la déforestation importée et de préservation de la biodiversité. L'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit en effet aucune action dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, alors que le secteur agricole et alimentaire représente le tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre. Au lendemain des accords de Paris, la politique alimentaire française doit prendre en compte la contrainte climatique pour pouvoir être intégrée à la stratégie de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui déjà, la politique agricole nationale se fonde sur quatre axes sociétaux : la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'ancrage territorial, la justice sociale et l'éducation. En 2016,

Depuis le début de son action, le Gouvernement a fait le choix d'une politique volontariste en matière environnementale et climatique, au niveau tant national qu'international. Ce combat pour la planète est au coeur de l'évolution de notre modèle productif

il n'est pas envisageable de cibler l'intégralité de cette politique sur ce seul enjeu. En effet, la politique alimentaire doit notamment permettre de lutter pour davantage de justice sociale, ou encore de mettre en valeur notre patrimoine alimentaire. Nous voterons donc contre l'amendement

L'article L. 3231-1 du code de la santé publique établit le programme national relatif à la nutrition et à la santé. Cependant, il ne fait pas mention des enjeux climatiques et environnementaux, alors que le secteur agricole et alimentaire est responsable du tiers des émissions françaises de gaz à effet de serre. La stratégie nationale bas carbone envisage une diminution radicale de ces émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, dans la perspective des engagements pris au travers

En outre, l'amendement tend à renforcer l'éducation à l'alimentation dans les programmes et les activités scolaires et universitaires : sessions sur la nutrition, la protection de l'environnement, la lutte contre la déforestation ou encore le bien-être animal. L'éducation à l'environnement est un enjeu essentiel de la formation des petits et des grands, et doit faire pleinement partie des formations en matière d'alimentation.

Par un courrier resté sans réponse, nous avons demandé au président de la commission des finances de revenir sur cette décision, qui frappe bien trop souvent nos amendements. L'amendement concerné visait à instaurer, entre autres dispositions, une obligation, pour la restauration collective publique, de proposer au moins 30 % de produits issus de l'agriculture biologique.

Nous considérons cette interprétation comme particulièrement hâtive et jugeons que la commission des finances n'a pas envisagé la mesure sous tous les angles. Cette obligation de recourir à hauteur de 30 % à des produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective ne saurait nécessairement induire une augmentation des charges publiques. peut tout à fait être envisagée à coût constant, voire à coût réduit. Tout d'abord, on peut ajuster la composition des menus, par exemple en supprimant un repas carné par semaine, comme cela sera proposé au cours du débat. Ensuite, on peut s'approvisionner en circuit court, notamment en vente directe, ce qui réduit considérablement les coûts d'approvisionnement. Une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire peut également permettre de substantielles économies de volume, et partant une réduction des achats de denrées alimentaires. Enfin, les municipalités peuvent accompagner cette démarche par la création de régies municipales agricoles, permettant une production locale de fruits et légumes à même d'approvisionner la restauration collective des établissements publics. C'est le cas de la commune de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, qui propose, dans les cantines de ses établissements publics, des menus 100 % bio pour un prix de revient par repas de 1,86 euro, défiant toute concurrence. Nous sommes bien loin des 8 euros que coûte en moyenne aux deniers publics chaque repas de cantine scolaire

nous avons la chance, en France, d'avoir un modèle alimentaire fort, probablement le plus remarquable qui soit. Néanmoins, depuis une trentaine d'années, progressivement, parfois insidieusement, ce modèle est remis en cause et fragilisé. Certes, le développement des magasins de grande surface, proposant des assortiments gigantesques de produits alimentaires, conjugué à un rythme de vie individuelle et familiale réduisant le temps de préparation des repas et le temps passé ensemble à table, a fortement influencé les choix alimentaires. On pourra arguer que l'industrialisation de la fabrication des produits alimentaires et l'allongement des circuits de distribution ont fait gagner en sécurité alimentaire, mais, il faut le dire, cela a souvent été au détriment de la valeur nutritionnelle et organoleptique des produits. La teneur des produits en sucres libres, c'est-à-dire sans valeur nutritionnelle, n'a cessé de progresser en trente Qui sait, par exemple, que la consommation de boissons sucrées a sextuplé dans le même temps et que celle des produits riches en glucides simples, tels que gâteaux ou crèmes glacées, a été multipliée par quatorze ? Cette exposition permanente au sucre est bien une réalité. ne cesse de produire ses effets délétères. Il faut de dix à quinze ans d'exposition à ces produits pour voir émerger toutes les maladies chroniques non transmissibles de notre monde moderne

des carottes râpées : on a perdu le bon sens le plus élémentaire ! L'enjeu est donc, monsieur le ministre, de prendre des mesures protectrices fortes et incitatives pour que l'industrie agroalimentaire incorpore beaucoup plus de matières agricoles à bien meilleure valeur

issus de circuits courts, répondant à des critères de développement durable. Je proposerai également de privilégier dans la restauration collective des produits issus des projets alimentaires territoriaux, et de supprimer la référence à la haute valeur environnementale de niveaux 1 et 2, pour ne retenir que le

Pourtant, depuis 2009, nous débattons de la fixation d'un taux de 20 % de produits issus de l'agriculture biologique pour l'approvisionnement de la restauration collective assurée par les personnes publiques. Même si la puissance publique ne peut pas agir directement et rapidement sur chaque assiette, la restauration collective constitue un point de départ. C'est là que nous pouvons faire découvrir ou favoriser une autre manière de se nourrir. Nous sommes déjà en retard. Depuis le 5 mai, la France vit pour cette année à crédit, alertent certaines associations. L'agriculture n'en est pas, tant s'en faut, seule responsable. Mais ce système d'élevage intensif que nous avons fait peser sur nos agriculteurs et que nous avons Nous devons favoriser les conversions vers l'agriculture biologique, dans le respect des êtres humains qui nous nourrissent et en leur garantissant un revenu décent. Nous devons favoriser une alimentation bio de qualité et, surtout, d'origine locale, parce que nous sommes confrontés à une situation critique. Notre nourriture a un impact sur notre santé, particulièrement sur celle de nos enfants.

la réponse à ma petite question, monsieur le ministre -qui affaiblissent nos normes sociales et environnementales, encouragent cette recherche de marges, de profits, et sont destructeurs pour la planète. Cet enjeu-là englobe

Je souhaite très vivement que nous n'opposions pas agriculture classique et agriculture biologique, mais que nous adoptions une démarche pragmatique pour permettre à nos agriculteurs de saisir toutes les opportunités locales, mais aussi pour répondre aux attentes du marché et de la société.

pour nos agriculteurs. J'y reviendrai, mais je pense qu'il n'est pas du rôle du Parlement de légiférer sur des questions scientifiques aussi spécifiques. La suppression des produits phytosanitaires

permet de ne pas ajouter des normes supplémentaires trop restrictives en matière de restauration collective. Je pense ici aux maires qui se trouvent confrontés aux difficultés liées à la restauration scolaire, par exemple, et aux difficultés d'approvisionnement. Dans nos territoires, les agriculteurs ont le souci de proposer des produits de qualité. Ce serait bien méconnaître les modes de production que d'imaginer que l'agriculture biologique pourrait permettre à elle seule de régler la question importante de l'accès à une alimentation saine.

Si je reste convaincue que le « manger local » doit être soutenu et encouragé, nous devons veiller à ne pas opposer les différentes filières. Elles constituent la formidable richesse de l'agriculture française les circuits courts sont un formidable levier économique pour créer de l'activité dans nos campagnes.

Mais nous souhaitions aller plus loin et fixer un cap ambitieux, en engageant les collectivités dans une démarche vertueuse. En effet, pour le dire schématiquement, 20 % de produits bio dans un repas, cela correspond à un morceau de pain et à un fruit : rien d'inaccessible Nous ne doutons pas une seconde que les établissements publics s'adapteront sans effort et que l'offre française de bio est largement suffisante pour répondre à cette nouvelle demande. Car le bio est un mode de production par essence local. Je profite de l'occasion pour battre en brèche l'argument fallacieux, trop souvent utilisé dans cet hémicycle, selon lequel le bio consommé en France viendrait de partout, sauf de France ! C'est parfaitement faux : selon le ministère, 69 % des aliments bio consommés en France sont produits en France. Aucune autre filière, aucun autre mode de production ne se peut se targuer d'être plus local que le bio. À titre de comparaison, dans la restauration française, de 50 % à 70 % de la viande produite de manière traditionnelle vient de l'étranger. C'est justement sur ce point que nos collègues de la majorité sénatoriale, fervents défenseurs de nos territoires, devraient nous rejoindre. Au-delà des considérations écologiques et sanitaires, le bio permet de revitaliser nos territoires, il crée deux fois plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle, il développe les circuits courts la vente directe et irrigue l'économie locale,

Il ne s'agit surtout pas, cela a été dit, d'opposer un type d'agriculture à un autre. Mais c'est une conviction que l'on ne nous ôtera pas et que ce débat renforce : le bio et les circuits courts sont les moyens les plus efficaces de parvenir à un revenu paysan décent, dans le respect de l'environnement. Il faut donc amplifier, favoriser, encourager le développement du bio et des circuits courts en France.

La parole est à Mme Angèle Préville, sur l'article. Monsieur le ministre, une alimentation saine, durable et accessible à tous, quel bel affichage ! Je le dis sans ironie. C'est ambitieux et alléchant, si je puis me permettre.

Nous verrons, lorsque la loi s'appliquera, si l'alimentation devient effectivement saine, durable et accessible à tous. Les consommateurs sont de mieux en mieux informés, se sentent de plus en plus concernés, s'impliquent comme jamais et font des choix. Le changement vient d'eux, vient de nous tous, consommateurs, et la tendance est là, forte, telle une lame de fond, portée en particulier par les jeunes couples avec enfants. Donc, l'avenir est là : le bio connaît une croissance à deux chiffres.

bon pour les agriculteurs, bon pour la santé, respectueux de l'environnement et de la biodiversité et, surtout, c'est bon dans l'assiette ! Notre gastronomie a été inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. C'est à nous, Français, qui avons hérité de ce patrimoine immatériel, de promouvoir une alimentation saine, durable, goûteuse,

que faisons-nous de tous ces additifs, de tous ces édulcorants, épaississants, émulsifiants, colorants et autres exhausteurs de goût ?

toute la société. Il faut lui donner une crédibilité et un modèle économique. Monsieur le ministre, affirmons une ambition forte à l'échéance de dix à quinze ans. Il y a de la place pour tout le monde : un tiers d'agriculture conventionnelle, un tiers d'agriculture à

obligation de résultat plutôt que des principes normatifs. Elle a été un peu expérimentée, mais insuffisamment. Un label de ce type pourrait rassurer

même si des stratégies d'achat intelligentes peuvent parfois permettre d'augmenter, en valeur comme en volume, la part du bio dans les approvisionnements, pour un certain nombre de produits, le différentiel de coût reste un handicap majeur.

et, à ce titre, j'ai assisté à la séance au cours de laquelle les services de l'État ont présenté les éléments de ce projet de loi, en particulier son futur article 11. Celui-ci devait introduire des normes ayant des conséquences financières pour les communes et les collectivités en général.

Enfin et surtout, les élus, maires, présidents de département, présidents de région, revendiquent leur responsabilité dans la mise en oeuvre du dispositif.

contre-productive pour favoriser l'utilisation des produits locaux en restauration collective. Une viande produite selon un cycle de production intensif et court importée par bateau pourrait ainsi être considérée comme plus « vertueuse » qu'un produit d'élevage extensif local. De plus, cette analyse est complexe, requiert beaucoup de données et peut être difficile à fournir pour un petit producteur. Le principe de circuit court respectant des critères de développement durable est ainsi bien plus opérant pour relocaliser l'alimentation et garantir un revenu aux producteurs. Dans le même esprit, je proposerai de favoriser l'approvisionnement des restaurants collectifs des projets alimentaires territoriaux garants d'une relocalisation efficace.

Des filières de commerce équitable locales qui répartissent la valeur se développent avec succès sur notre territoire. Pourquoi ne pas prévoir de favoriser l'inclusion de leurs produits dans la restauration collective ? Je ne comprends pas la référence à la loi de 2005, et je propose de qui avait été introduite à l'Assemblée nationale. Enfin, cet amendement supprime la référence aux données sous certificat de conformité des produits, de même que celle aux produits de haute valeur environnementale et 2, qui ne présentent pas de garanties suffisantes de qualité, surtout au regard des autres produits cités dans l'article. Cette rédaction me paraît satisfaisante pour garantir l'objectif de relocalisation et de qualité de l'approvisionnement en restauration collective,

à reprendre les objectifs de composition des menus avec 50 % de produits répondant à des exigences de qualité, dont 20 % issus de l'agriculture biologique.

Les produits labellisés « régions ultrapériphériques » sont ajoutés. Le seuil au-delà duquel un plan pluriannuel de diversification des protéines doit être élaboré est relevé de deux cents à trois cents couverts par jour en moyenne. L'information et la consultation régulières des usagers sont réintroduites et étendues aux établissements de santé, sociaux, médico-sociaux et pénitentiaires, qui avaient été oubliés, mais les gestionnaires seront les seuls juges des moyens à mettre en oeuvre.

de l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité

par l'article 11 aux seuls gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration scolaire et universitaire, des crèches, des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires, ce qui veut dire que les services de restauration publique destinés aux agents administratifs, les casernes par exemple, seront exclus. Or je considère qu'il n'y a pas lieu de mettre de côté un pan entier du service public. Vous proposez de préciser que les objectifs de 50 % et de 20 % peuvent être dépassés,

son champ est plus restreint que celui que nous proposions à travers notre amendement, puisqu'il ne prend pas en compte la restauration publique administrative. Or, vous le savez, nombre de nos

de Mme Loisier ne va pas aussi loin que l'on pourrait le souhaiter, car il tend à restreindre un certain nombre de champs, notamment sur la question des régions ultrapériphériques,